des opérations subventionnées à hauteur en moyenne de 149 000 euros. Les opérations les plus coûteuses, bénéficiant de fortes subventions, absorbent une part importante de l'enveloppe de la DETR, même si les pratiques varient d'un département à l'autre. À titre de comparaison, le montant moyen des subventions attribuées à la demande des sénateurs au titre de feu la réserve parlementaire était de 6 788 euros en 2017 et le coût total moyen des projets subventionnés, de 102 000 euros. Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement prévoit de réserver une part de 15 minimum de l'enveloppe départementale de DETR aux projets dont le coût n'excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient alors attribuées par le préfet de département.

Avec un niveau record de 87 millions de visiteurs internationaux, la France a confirmé en 2017 sa première place de destination la plus visitée au monde.

selon Atout France, et 2 millions d'emplois directs et indirects selon le Gouvernement. Renforcer l'attractivité des destinations françaises nécessite une politique d'investissement ambitieuse pour les communes touristiques ; il est donc indispensable que la DSIL permette de soutenir les projets des communes.

comme la rénovation des bâtiments scolaires, la transition énergétique, la construction de logements. À trop vouloir élargir ses missions, nous risquons de la vider de son contenu.

le ministre, le rédacteur de cet amendement, que nous soutenons largement, souhaitait mettre en avant l'importance, pour l'ensemble des communes, y compris rurales, de travailler sur l'investissement touristique, qui est un facteur de progrès et de création d'emplois.

et la vôtre, monsieur le ministre, concernant les projets éligibles à la DSIL. Il est vrai que nous faisons partie de la commission DETR. Celle du département des Ardennes, que vous connaissez relativement bien,

de subventions est contraire aux principes de la décentralisation. Une réelle concertation serait à tout le moins nécessaire avant d'envisager une réforme de la DGE. Afin d'éviter toute difficulté dans la répartition de cette dotation, le présent amendement prévoit seulement que les sommes nécessaires pour honorer la garantie selon laquelle l'attribution d'un département au titre de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente sont prélevées, si nécessaire, sur la part principale

des départements. Je n'ai pas d'opposition de principe à la réforme proposée de la DGE. S'il ne s'agit plus d'un taux de concours sur les dépenses d'aménagement foncier, une part de cette nouvelle dotation de soutien est

du code général des collectivités territoriales, que les syndicats d'énergie mentionnés dans le code mettent en oeuvre depuis de nombreuses années pour financer des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière d'éclairage public et de transition énergétique. Toutefois, certaines préfectures- direction générale des collectivités locales, la DGCL -ont récemment estimé que ce dispositif pouvait uniquement être utilisé pour financer des dépenses de fonctionnement ou d'investissement sur des équipements directement liés à l'exercice de la compétence de distribution d'électricité, ce qui exclut par conséquent les actions que je viens d'évoquer, notamment sur les réseaux d'éclairage public, qui ne font pas partie,

Ces amendements visent à permettre aux syndicats d'énergie de continuer à percevoir des fonds de concours de communes pour financer pour leur compte des travaux en matière d'éclairage public et de transition énergétique, alors que certaines préfectures

numérique pour les personnes morales. En l'état actuel du droit, les collectivités sont obligées de mettre en place des dispositifs pour le paiement dématérialisé des personnes morales, tout en étant contraintes de conserver

Toutefois, la population prise en compte dans le calcul de la DETR départementale est la population des communes de moins de 20 000 habitants appartenant à des EPCI de moins de 75 000 habitants. Ces critères cumulatifs excluent d'emblée du mode de calcul de la DETR toutes les communes rurales appartenant à des intercommunalités de plus de 75 000 habitants. Le paradoxe est que les communes rattachées à des EPCI de plus grande taille, à la suite des différentes réformes de la carte intercommunale voulue par les gouvernements successifs, continuent en très grande majorité à être éligibles à la DETR, compte tenu de leur faible potentiel financier, mais ne sont plus prises en compte pour le calcul de l'enveloppe départementale. Les collectivités sont donc sanctionnées au regard de leur effort de rationalisation de la carte intercommunale. Cette proposition revient simplement à faire correspondre la base servant de calcul à la DETR avec les populations des communes effectivement éligibles dans un département donné. Il ne s'agit nullement de remettre en cause les critères d'éligibilité à la DETR, mais de revenir sur le mode de calcul de la répartition départementale pour ne pas défavoriser les communes, notamment rurales, qui, sous l'impulsion des dernières politiques, se sont regroupées au sein de grands EPCI.

aurait pu prendre l'exemple de sa commune de 3 000 habitants dans le Nord, qui a toujours été éligible à la DETR jusqu'en 2014, parce qu'elle était rattachée à un EPCI de petite taille. La population de sa commune était donc à l'époque prise en compte pour le calcul de l'enveloppe départementale. À présent qu'elle a rejoint une communauté d'agglomération beaucoup plus large, qui compte 159 000 habitants, la population de sa commune n'est plus prise en compte pour le calcul de la dotation. Le Gouvernement a d'ailleurs lui-même reconnu ce paradoxe, en faisant adopter un amendement à l'Assemblée nationale permettant aux EPCI de plus de 75 000 habitants d'être désormais éligibles à la DETR, sous certaines réserves. Quel est l'avis de la commission ? Cet

Parmi les raisons qui me font plaider pour une métropole du Grand Paris véritablement intégrée, qui supprimerait les départements de la petite couronne et celui de Paris, il y a bien cette raison-là.

composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen

défavorable.

le Sénat va maintenant statuer, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, sur les articles qui portent récapitulation de ces crédits.

des votes qui sont intervenus lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances. Je mets aux voix l'ensemble constitué de l'article 39 et de l'état B annexé. Je mets aux

Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les plafonds d'emplois ministériels du transfert du contentieux social aux futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance. Ainsi, il est proposé d'augmenter de 22 équivalents temps le plafond d'emplois du ministère de la justice et de réduire de 5 ETP celui du ministère des solidarités et de la santé. L'augmentation totale du plafond des emplois de l'État est par conséquent de 17. La contrepartie en crédits de ces mouvements était prévue par les amendements nII-435 et II-436, respectivement adoptés dans le cadre de l'examen des missions « Solidarité, insertion et égalité des chances » et « Justice ». Quel

Le plafonnement d'emplois pour les établissements à autonomie financière à l'étranger est un principe qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il avait été introduit par Michel Charasse et Adrien Gouteyron, avec le soutien de la commission des finances du Sénat, dans la loi de finances pour 2009.

Cette ressource d'emplois n'apparaît donc pas comme une nécessité prégnante. Par ailleurs, je rappelle que le soutien au réseau culturel a été renouvelé en 2019, avec une stabilisation des moyens et la mise en oeuvre des annonces présidentielles visant à la création de dix alliances françaises par an, ou encore au renforcement du rôle de l'institut français en tant qu'opérateur de la promotion et de la diffusion du français dans le monde. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

messieurs les sénateurs, l'article 15 de la LOLF prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. L'article 47 du PLF pour 2019 fixe la liste des programmes bénéficiant d'une telle exception. Cet amendement vise à l'élargir à trois programmes : le programme « Affaires maritimes », de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », compte tenu du report de crédits pour lequel un besoin de 2019 est avéré le programme « Soutien à la politique de l'éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire », compte tenu du calendrier d'opérations immobilières ; enfin, le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission « Justice », compte tenu du décalage de dépenses du Grand Plan d'investissement.

quelle est votre estimation des reports en 2018, et le décalage par rapport à l'année dernière, ce qui nous donnera le décalage sur le déficit public ?

aux voix l'article 47, modifié. Nous avons achevé l'examen des crédits portant récapitulation des crédits. Nous abordons maintenant l'examen des articles non rattachés.

est l'avis du Gouvernement ? En réalité, cette différence de traitement est liée au fait qu'il y a une réciprocité au sein de l'Union européenne.

je le rappelle, lorsqu'elle implique deux pays, c'est d'exiger soit une réciprocité, soit des mesures un peu plus restrictives. Au surplus, tel qu'il est rédigé, votre amendement va bien au-delà de l'exposé des motifs que vous présentez puisqu'il fait bénéficier

Cette création d'un nouvel étage dans la lutte contre la fraude fiscale va dans le bon sens en intégrant que l'administration pourra agir lorsqu'un montage sera « principalement » fiscal. Cela veut dire que l'entreprise devra démontrer la nature économique du montage dont l'administration juge qu'il a « principalement » un but d'optimisation fiscale. Si nous réfléchissons un peu, il devrait être naturel qu'une entreprise ne s'organise qu'avec un objectif de nature économique, mais nous savons tous que tel n'est pas le cas ! C'est la fameuse « zone grise » entre optimisation fiscale et fraude fiscale je regrette qu'un amendement ait retardé d'une année l'application de cette disposition, qui émane pourtant d'une directive européenne. Faudrait-il laisser du temps aux entreprises pour faire le ménage, plutôt que de donner toute latitude à l'administration pour qu'elle lutte contre la fraude, qu'elle la réprime et récupère

Je vous rappelle que le Sénat a adopté une proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise. Ce texte traduisait notamment la volonté de faciliter la reprise interne en abaissant le nombre minimum de salariés repreneurs requis

afin de favoriser l'utilisation d'un dispositif qui permet de sauvegarder des emplois sans susciter d'effets induits négatifs, un an d'ancienneté permettant de se prémunir contre d'éventuels contrats de complaisance.

prévu dans le cadre du crédit vendeur n'a été utilisé que dans deux cas en 2017, pour un montant d'impôt sur le revenu total inférieur à 300 000 euros. Les différents assouplissements proposés au présent article pourraient toutefois ne pas suffire pour relancer le crédit vendeur, dans la mesure où il n'apporte aucune solution à la double peine dont est victime le cédant en cas de défaut de paiement du cessionnaire. Nous avons le sentiment de passer, en fait, d'une mesure quasi inappliquée à une mesure fort hypothétiquement mise en oeuvre

n° II-940 rectifié. L'article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d'élargir l'éligibilité à l'étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d'un crédit vendeur aux cessions d'entreprises individuelles ou de sociétés. Son objectif est de faciliter le développement du crédit vendeur qui permet au repreneur d'acquérir l'entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. Or ce recours au crédit vendeur est, certes, élargi par le présent texte, mais demeure limité aux entreprises employant moins de cinquante salariés et dégageant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros.

ou, en tout cas, à mettre en place un nouvel impôt sur le patrimoine. Ce rétablissement s'impose aujourd'hui, au nom de la justice fiscale que nos concitoyens appellent clairement de leurs voeux. La suppression de cette imposition a en effet constitué un cadeau fiscal inespéré pour les plus riches. L'étude menée par l'Institut des politiques publiques est, à cet égard, extrêmement claire : le pouvoir d'achat des 1 % les plus aisés de nos concitoyens a crû de 6 % depuis un an.

de nos concitoyens de plus de 3 milliards d'euros, soit 0,2 point de revenu disponible brut. Par ailleurs, aucun élément ne vient confirmer que la suppression de l'ISF ait mené à plus d'investissement dans nos entreprises ou encore à plus de créations d'emplois. Avec la, le Gouvernement a encore renoncé à près de 4 milliards d'euros de recettes fiscales afin de favoriser le pouvoir d'achat de quelques-uns. Pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus modestes ne cesse, lui, de se dégrader Nous appelons donc à une répartition plus équitable de l'effort fiscal ; nous demandons le rétablissement de l'ISF et la suppression de la, ainsi que le retrait de l'article 51

aviez par ailleurs- « en même temps » -, considérablement augmenté la fiscalité sur les carburants, qui devait peser de façon accrue sur nos concitoyens les plus modestes.

Par cette disposition, le Gouvernement ouvre en effet la voie à tous les abus et encourage l'optimisation fiscale. Pour rappel, une récente étude menée par trois chercheurs, parmi lesquels le chercheur français Gabriel Zucman,

le Gouvernement permet donc aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France de ne pas être imposés sur les plus-values qu'ils réaliseront s'ils cèdent leurs titres et participations deux ans après avoir quitté la France. Ce délai de deux ans n'est pas suffisant, et le délai de cinq ans proposé pour les patrimoines de plus de 2,57 millions ne l'est pas plus : il est en effet trop facile de s'installer pendant deux ans dans un pays à faible fiscalité afin de liquider ses actions La majorité présidentielle fait encore une fois un cadeau aux contribuables français les plus riches, alors que nos concitoyens les plus modestes, qui étaient déjà censés subir la hausse de la fiscalité du carburant, vont de toute manière endurer la sous-indexation des pensions de retraite et de plusieurs prestations sociales. Encore un exemple d'injustice fiscale ! La situation sociale exige la suppression de cet article.

alléger les contraintes du droit du travail : on connaît cela par coeur ! Ce nouveau dispositif cible les cessions effectuées deux ans après le départ de France pour éviter les comportements d'optimisation consistant à faire un aller-retour de courte durée à l'étranger pour réaliser sa plus-value. Cela rappelle curieusement le mécanisme des « » : dans cet arbitrage de dividendes, on se déleste pendant deux jours

matière d'impôt. Nous avons obtenu l'accord de l'Allemagne ! Je ne crois pas avoir vu un gouvernement se saisir de ce sujet avant nous, alors que d'autres étaient en position de le faire ces dernières années. avancées majeures en matière de convergence fiscale, dans le cadre des futures directives ACIS et ACCIS, afin de limiter les effets du fiscal en Europe. la fraude, qu'a défendue M. Darmanin, a renforcé les dispositifs internes de lutte contre la fraude : aggravation des sanctions, création d'une police fiscale, publicité des sanctions fiscales pour les fraudes graves, enfin fermeture du guichet de régularisation pour les Français ayant des comptes non déclarés à l'étranger.

Mais Mme May ne va pas se laisser faire : vous pensez bien qu'elle a déjà sorti de son chapeau les arguments nécessaires pour les retenir. Elle avait déclaré, au lendemain du vote pour le Brexit : « Je vais faire en sorte que le Royaume-Uni devienne le meilleur endroit au monde pour faire du . » Alors, bon courage

La réforme envisagée aujourd'hui n'a pas pour objectif de supprimer cette taxe, mais simplement de l'aménager et de tenir compte du fait que tous les Français qui partent de France ne le font pas pour des raisons fiscales.

Les contribuables se trouvent dans la situation suivante : l'a pour effet de leur faire payer l'impôt sur la plus-value dès qu'ils partent de France, alors qu'ils n'ont pas vendu les actifs concernés. C'est la raison pour laquelle ils bénéficient, de la part de l'administration fiscale, d'un sursis de paiement qu'ils doivent garantir par des cautions bancaires.

s'il parvient à démontrer que le changement de domicile n'avait pas un but principalement fiscal. La formule utilisée à l'article 167 du code général des impôts- « avec pour motif principal d'éluder l'impôt » -est source d'insécurité juridique. Déterminer à l'avance si le motif principal d'une donation est fiscal s'avère extrêmement compliqué et, surtout, subjectif. Or le droit se doit d'être objectif

Or cette définition de l'abus de droit, fondée sur le « principalement fiscal », a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elle avait « pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ». Pour autant, l'article 167 du code général des impôts n'a pas été modifié. Je propose donc, simplement, de corriger cette faiblesse en revenant à l'ancienne rédaction, donc au motif « exclusivement fiscal », qui est beaucoup plus facile à appréhender. Quel

qui sont domiciliés dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Il nous semble donc que l'exigence ici contestée ne s'appliquerait à l'avenir qu'aux cas de domiciliation dans des territoires dont

ce jour, l'impôt établi à l'occasion du transfert du domicile fiscal hors de France fait l'objet d'un dégrèvement d'office ou d'une restitution. C'est notamment possible lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, ou en cas de décès du contribuable et si les titres ou créances constatés lors du transfert demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du décès, du décès, ou encore pour les plus-values latentes, à l'expiration d'un délai de conservation des titres de quinze ans suivant le transfert du domicile fiscal, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai. L'article 51 affaiblit donc très fortement la portée de l', alors qu'il s'agit d'un dispositif anti-abus en matière d'exil fiscal, qui a rapporté près de 138 millions d'euros entre 2012 et 2017 et dont les impositions restant en sursis de paiement s'élevaient à 5,3 milliards d'euros au mois de décembre 2017. C'est pourquoi il est proposé, en cohérence avec les travaux réalisés lors de l'examen du projet de loi relative à la lutte contre la fraude, de renforcer les conditions du nouveau dispositif.

finances, mais uniquement pour les patrimoines mobiliers les plus importants, conservant le délai de deux ans pour les autres patrimoines. La création d'un nouveau seuil de patrimoine pourrait entraîner une véritable insécurité juridique, car la valorisation des titres d'une société est un exercice complexe, source de contentieux importants entre les contribuables et l'administration fiscale. C'est pourquoi il est proposé de simplifier, afin d'éviter cette insécurité juridique, en passant le délai de conservation à cinq ans, quelle que soit la nature

le régime des plus-values immobilières, qui, aujourd'hui, est un régime dégressif sur vingt-deux et trente ans, en fonction soit de la plus-value, soit du prélèvement social, avec un taux très élevé : 36,2 %.

Travaillons au présent et dans un futur immédiat pour aboutir

mais nous sommes impatients de voir ce que le Gouvernement nous proposera pour essayer de rectifier le tir. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, les DMTO sont en train de s'effondrer-

à préciser les données statistiques devant figurer au sein du futur document de politique transversale. J'en comprends l'objectif, à savoir ne pas oublier certaines données, mais je ne suis pas certaine que la loi doive entrer dans ce degré de détail. J'ajoute que, paradoxalement, cette liste limite le contenu du document, alors qu'il convient de conserver une certaine souplesse. messieurs les sénateurs, je m'engage à ce que mes services fournissent les données les plus complètes possible en fonction des capacités de restitution statistique des applications et en prenant bien en compte les éléments présentés dans ce sous-amendement. La parole est à M. le rapporteur général.

d'évaluer le manque à gagner pour les finances publiques d'une définition trop favorable d'un établissement stable, particulièrement pour les entreprises du numérique, dans les conventions fiscales actuellement en vigueur. Cette demande s'appuie sur les récentes décisions de justice et les dernières préconisations de l'OCDE et de la Commission européenne. il s'agit de tenir compte de la décision du tribunal administratif de Paris dans l'affaire qui a opposé l'État à la société Google selon laquelle les termes de la convention fiscale franco-irlandaise ne permettent pas à l'État français, du fait de l'absence d'établissement stable, de réclamer les impôts sur les sociétés calculés par la DGFiP-

à l'établissement stable. Lorsque la convention multilatérale de l'OCDE ne permet pas une telle évolution, parce que l'autre État n'a pas souhaité la mettre en oeuvre, ce qui arrive, la France s'attache à promouvoir ces nouveaux standards dans un cadre bilatéral, tout en travaillant activement à une réforme de l'imposition des activités numériques au sein de l'Union européenne et de l'OCDE.